La séance est reprise. Mes chers collègues, en accord avec le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants, la nomination des membres de la mission d'information sur les influences étatiques extra-européennes dans le monde

au bon moment- je pense, comme mon collègue Jacquin, qu'il faut cesser de procrastiner -, qui puisse jouer un rôle moteur pour le report modal et qui ne réduise pas les capacités des transporteurs à réussir la transition de la décarbonation. Nous proposons donc un dispositif national, ce qui éviterait les effets de bord, les concurrences entre régions, le poids excessif des coûts de collecte et l'illisibilité pour les usagers. une taxe kilométrique plutôt progressive, destinée surtout à avoir un impact sur les trajets longs, pour lesquels l'offre ferroviaire, qui doit doubler d'ici à 2030, est principalement destinée. d'un accompagnement des transporteurs, de façon à leur assurer la répercussion du coût sur les chargeurs, sous forme de bas de page obligatoires sur les factures. Il s'agit de leur garantir que ce n'est pas leur marge qui sera ponctionnée par cette contribution. Enfin, nous proposons un fléchage des recettes vers la transition du transport de marchandises et les investissements nécessaires.

le difficile équilibre entre, d'une part, la volonté d'améliorer un dispositif aux effets pervers nombreux, et, d'autre part, la nécessité de faire contribuer le secteur du transport routier de marchandises

nous voterons cet amendement, même si nous avons déposé un amendement assez proche, placé après l'article 32. Nous n'avons pas le temps de débattre, mais vous voulez prendre le temps

donc un avis défavorable.

dont le développement significatif dans les régions touristiques crée un fort surtrafic, notamment en raison du non-respect de la réglementation en vigueur. Ce type de tourisme, dont la trajectoire est ascendante et qui a été renforcé par l'épisode de la crise sanitaire, n'est pas sans impact sur des écosystèmes fragiles, puisque la pratique d'incivilités écologiques, comme le camping sauvage, reste, hélas, répandue. La crise sanitaire a d'ailleurs mis en exergue les conséquences chaotiques auxquelles certains territoires ont été confrontés face à l'afflux de ce mode de transport : sur-concentration, stationnement anarchique, camping sauvage, incivilités écologiques, etc. Dans le cas de la Corse, l'amplitude du phénomène est particulièrement notable, avec une moyenne annuelle de 28 000 entrées de camping-cars, concentrées sur une saisonnalité étroite et sur un relief marqué par des routes étroites et sinueuses. Certaines zones demeurent peu adaptées à ce type de véhicules, dont l'afflux massif, couplé au non-respect des règles de stationnement aux emplacements dédiés, accentue fortement le surtrafic routier, ainsi que les conflits d'usage. Lesdits amendements tendent donc à réguler cette pratique, en la conciliant avec le respect des impératifs écologiques particulièrement prégnants dans certaines régions, une fiscalité incitative au développement de pratiques vertueuses et durables.

que le bilan sur la trajectoire de décarbonation du transport routier de marchandises et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir doivent porter spécifiquement sur un type de véhicule

L'objet de cet amendement est de prévoir que la contribution assise sur le transport routier de marchandises, dont le présent article envisage la création, soit réduite pour les véhicules à faibles émissions. Plutôt que de prévoir une approche punitive, il s'agit exclusivement de stimuler l'émergence des marchés de véhicules lourds propres. Dans cette perspective, toute taxation devrait être différenciée en fonction du degré de pollution générée par le véhicule utilisé.

semble donc particulièrement opportun, toujours dans l'éventualité où, en 2028, le secteur n'aurait pas significativement réduit ses émissions.

puis la loi dite « Grenelle I » de 2009, avant la suspension, puis l'abandon, de ce qui était alors l'écotaxe. Le cas de l'Alsace est intéressant. En discussion depuis plus de quinze ans, la mise en place d'une taxe kilométrique deviendra réalité, à la suite de la publication de l'ordonnance du 26 mai 2021. Dès lors, le présent article prévoyait d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance, afin de permettre aux régions d'instituer des contributions spécifiques assises sur le transport routier de marchandises. Toutefois, la commission a estimé que cet article, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, soulevait un certain nombre d'interrogations, qu'il s'agisse d'un transfert de certaines voies du réseau national non concédé aux régions, est prévu par le projet de loi 4D, ou encore du calendrier, lequel paraît peu pertinent par rapport à la réforme en cours de la directive Eurovignette. Enfin, une zone d'ombre subsistait quant aux effets de bord, qui sont d'ailleurs, par exemple en Alsace, à l'origine d'une écotaxe régionale, mais qui se répercute de nouveau dans les départements limitrophes aux régions qui choisiraient de mettre en place d'une telle écotaxe. Nous avons une ambition- réussir la transition -et nous avons des atouts notre expertise, nos champions et notre expérience ferroviaire. Nous proposons, dès lors, une méthode : favoriser le report modal. La parole

à mettre en place un plan de hiérarchisation de la voirie, afin d'abaisser la vitesse de 50 à 30 kilomètres à l'heure au coeur de nos agglomérations. Ce dispositif existe déjà dans plusieurs centaines de villages et de villes, et il bénéficie en premier lieu aux personnes les plus vulnérables. L'Observatoire des mobilités émergentes

de conditionner l'opportunité de mettre en place une contribution sur le transport routier de marchandises à la non-réalisation d'une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre par le secteur d'ici à 2028. Cet amendement vise à prévoir une redevance, comme le permet la directive Eurovignette 3, qui autorise les États à introduire dans les péages routiers des poids lourds une prise en compte de coûts externes concernant la pollution de l'air et le bruit. le produit de cette redevance serait de l'ordre de 130 millions d'euros, un montant très éloigné des impacts financiers des externalités des transports. Mais l'introduction de ce principe pourrait avoir comme avantage de commencer à permettre la prise en compte des externalités dans les redevances d'utilisation des infrastructures de transport.

applicable aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes. Seraient donc également concernés les grands véhicules utilitaires légers, les VUL, dont le poids total autorisé en charge se situe entre 2,5 et 3,5 tonnes. Comme le souligne le rapport sénatorial de Nicole Bonnefoy et Rémy Pointereau, réalisé au nom de la mission d'information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux publié en mai dernier, le parc de ces VUL n'a cessé de croître ces dernières années pour constituer aujourd'hui la moitié du parc. Or ceux-ci sont de plus en plus utilisés pour le transport de fret et concurrencent ainsi les poids lourds, y compris sur les longues distances. Comme le soulignent les auteurs du rapport d'information précité, « les VUL sont soumis à une réglementation plus souple que les poids lourds ». Leur essor participe dès lors à la déréglementation, notamment sociale, du secteur par contournement des règles qui s'appliquent uniquement aux poids lourds. Il n'y a aucune raison qu'ils échappent, dès lors, à une redevance poids lourds qui, dans le cas contraire, accroîtrait encore la concurrence déloyale qu'exerce sur le secteur ce type de véhicule. L'amendement

les véhicules de charge supérieure ou égale à 3,5 tonnes. Dans un contexte où le transport de marchandises routier présente un bilan carbone très problématique, il s'agit d'encourager à la limitation de ce mode de transport entraînant des émissions de gaz à effet de serre élevées, selon le principe pollueur-payeur. Cela participe de l'encouragement au report modal vers le transport ferroviaire ou fluvial que portent les sénateurs socialistes depuis plusieurs années. Le choix d'une redevance kilométrique plutôt que d'une redevance permet de tenir compte de la pollution générée et de l'énergie consommée lors des trajets de longue distance. cet amendement a pour objet d'encourager les transports de courte distance, présentant des conséquences moindres en termes de consommation énergétique. à associer les conseils régionaux à la définition des axes et des sections de ces axes pour lesquels cette redevance serait demandée. Il s'agit d'une mesure cohérente avec la volonté du Gouvernement de transférer une partie des routes nationales aux régions, dans le cadre du projet de loi 3DS.

Le transport de marchandises routier représente un bilan carbone problématique. Il entraîne aussi, sur les axes qu'il emprunte, de nombreuses difficultés, notamment la saturation des voies et leur dégradation rapide. Ce dernier phénomène constitue une véritable problématique pour les finances publiques, alors même que l'État et les collectivités connaissent les plus grandes difficultés à entretenir le réseau existant. Une telle ressource permettrait de résoudre en partie cette difficulté. De nombreux pays étrangers, dont les voisins directs de la France, ont déjà instauré des « écotaxes », causant ainsi un report du trafic des camions étrangers sur les axes routiers Afin d'anticiper les mécanismes de déport consécutifs à l'instauration de taxes sur des portions isolées de territoires, sans cohérence avec l'ensemble du réseau routier régional, il est proposé que, au sein d'une même région, une taxe sur les poids lourds ne puisse être délibérée sans avis conforme des autres départements de cette

Mme Sabine Drexler. L'amendement n° 283 rectifié a pour objectif d'autoriser les régions à instaurer une redevance poids lourds. Or cette compétence relève désormais, en Alsace, de la Collectivité européenne d'Alsace, la CEA, créée en janvier dernier, qui fusionne les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Je voudrais rappeler ici la loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la CEA, qui transfère à celle-ci les routes et les autoroutes non concédées du domaine national et lui donne la possibilité de mettre en place une écotaxe sur ses axes routiers. Cette écotaxe, les Alsaciens l'attendent avec impatience, car notre territoire subit un trafic poids lourds très important sur l'A35 depuis 2005, date de la mise en place d'une taxe poids lourds en Allemagne. Depuis cette date, nous connaissons un report de circulation important, avec près de 3 000 poids lourds supplémentaires par jour. Nous subissons une augmentation très notable de la pollution de l'air, une pollution sonore, l'usure prématurée de nos infrastructures, des embouteillages quotidiens et une accidentologie élevée depuis plus de quinze ans. Les élus alsaciens sont, depuis lors, mobilisés pour mettre en oeuvre cette écotaxe. Dès 2005, le député alsacien Yves Bur avait déposé un amendement pour l'instaurer chez nous, ce qui avait d'ailleurs entraîné le projet de création d'une écotaxe nationale, abandonné en 2013 par le gouvernement socialiste.

Cela avait été négocié et voté au Parlement en 2019, et l'ordonnance du 26 mai 2021 fixe le cadre de sa mise en oeuvre. Le projet est donc en cours. Il aboutira en 2024, bien avant la limite de 2028 fixée par le texte.

Cette mesure est présentée comme cohérente avec le transfert à la CEA de la compétence des routes et autoroutes nationales non concédées, transfert qui a été voté en 2019. À l'époque, le Sénat avait voulu permettre aux départements lorrains d'instaurer cette taxe, mais l'Assemblée nationale et le Gouvernement avaient rejeté cette proposition de bon sens. L'autoroute A35 traversant l'Alsace est aujourd'hui saturée par le report des flux de camions en transit international, qui évitent ainsi les écotaxes poids lourds mises en place à l'étranger. Mais le Gouvernement refuse toujours de prendre en compte le phénomène de déport des camions sur les axes départementaux voisins de l'Alsace, qui, eux, ne disposent pas de la faculté de mettre en place une redevance. Les routiers qui voudront échapper à l'écotaxe feront donc un détour par l'A31, en Moselle et en Meurthe-et-Moselle, pour rejoindre la France. Cette autoroute est connue pour être déjà saturée par un trafic structurel de marchandises, occasionnant de nombreux embouteillages et une dégradation rapide du réseau 10 000 à 15 000 camions transitent quotidiennement par la Lorraine. Pour les mêmes raisons qui ont poussé le Gouvernement à prévoir une écotaxe en faveur de l'Alsace, et par souci de justice et d'équilibre entre les départements du Grand Est, il est proposé de donner à la région Grand Est la faculté d'instaurer une redevance sur l'ensemble des départements la composant. La

Cela a été dit, les Alsaciens attendent cette mesure depuis de nombreuses années et, dans les faits, elle est déjà en train de se mettre en place. Il s'agit donc d'un sous-amendement cohérent : notre projet d'écotaxe avance et sera effectif dès 2024, sans que l'on ait à attendre que d'autres territoires se positionnent. Nous comprenons bien les préoccupations de nos collègues des territoires voisins, mais les Alsaciens ont pris leur destin en main sur ce dossier et ne peuvent plus attendre, une nouvelle fois, que d'autres collectivités trouvent les moyens de mettre en oeuvre de leur propre écotaxe. Nous invitons d'ailleurs nos collègues du Grand Est à s'émanciper, eux aussi, sur ce sujet.

sous-amendement de cohérence, qui vise à harmoniser les compétences entre la région Grand Est et la Collectivité européenne d'Alsace, sans pour autant s'opposer à ce qu'une écotaxe similaire puisse être mise en place dans d'autres territoires. Il s'agit donc de préciser que la CEA conserve la pleine souveraineté pour l'instauration d'une écotaxe sur son domaine public et d'éviter que les usagers des autoroutes alsaciennes ne soient redevables de deux taxes du seul fait de l'utilisation de ces voies. L'amendement n° 1859 rectifié

corridor parallèle à celui du Rhin. Ne nous dites pas que cet amendement tendrait à menacer l'équilibre politique : nous sommes dans la cohérence du texte voté à l'unanimité

Sans en remettre en cause le bien-fondé, ce sous-amendement vise, par cohérence, à harmoniser les compétences entre la région Grand Est et la CEA.

de l'écotaxe. Lors de l'examen de l'article 32 en commission, nous avons fait le choix de responsabilité de ne pas adopter un amendement de suppression ou de rejeter la responsabilité de cette mesure sur le projet de loi 4D. Cependant, il nous a paru indispensable de revoir un dispositif au périmètre flou aux effets pervers nombreux, par lequel le Gouvernement s'en remettait aux régions pour ne pas endosser la responsabilité de la mise en place une écotaxe. Ces amendements visent à mettre en oeuvre à courte échéance un dispositif autrement plus contraignant et qui n'est pas

dans la CEA illustre les périls du dispositif envisagé. Quels seront, demain, les effets de bord sur les départements et régions limitrophes ? Si le dispositif prévu empêche le report modal de camions étrangers effectuant du transit, il risque de susciter des effets de bord des transporteurs français, qui se décaleront peut-être sur les régions limitrophes. La position de cette assemblée doit être claire : nous devons nous opposer à la mise en place, dès demain, d'une nouvelle écotaxe qui ne serait ni discutée ni maîtrisée et qui provoquerait une concurrence fiscale entre les différents territoires.

À ce jour, les camions venant du nord de l'Allemagne traversent l'Alsace- vous le savez, vous le vivez depuis 2005, depuis la mise en place de la la taxe allemande sur les camions -, afin de profiter des 200 kilomètres d'autoroutes gratuites.

procède d'une volonté partagée de compléter la contribution poids lourds de la CEA par une protection du sillon lorrain contre un dommage collatéral évident. Il est temps de désamorcer les logiques de ressentiment ou d'égoïsme qui montent dans ce Grand Est, lequel a si peu rencontré l'adhésion des électeurs dimanche dernier.

européens qui traversent ces zones, et le risque de report a été estimé à près de 4 000 véhicules par jour sur l'A31, qui est l'une des autoroutes les plus encombrées de France. Au nord de Metz, on est à plus de 100 000 véhicules par jour, avec près de 11 000 poids lourds,

je l'assume ! Franchement, il y a beaucoup de politique, ces temps-ci, avec cette ordonnance sur l'Alsace qui a été présentée quelques jours avant les élections régionales, alors que la ministre Klinkert, qui la défend, est aujourd'hui en campagne, sans étiquette. M. Rottner, me dites-vous,

par une foultitude de cosignataires, comme l'a aimablement et intelligemment relevé mon collègue Jacques Fernique.

territoire. Nous en avons suffisamment parlé ; vous nous avez dit que le Gouvernement ne pouvait pas mettre en place des écotaxes régionales et donner cette responsabilité aux régions et qu'il fallait une cohérence en

Le montant des recettes générées par cette augmentation permettrait de financer davantage, d'une part, l'amélioration des infrastructures de transport, en abondant l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, l'Afitf, et, d'autre part, le développement du ferroviaire, en compensant une partie du déficit des trains d'équilibre du territoire. Pour ne pas pénaliser les circuits courts et les transporteurs locaux et cibler prioritairement les longs trajets, pour lesquels le fret routier ou fluvial est plus pertinent, la taxe ne s'appliquerait qu'à partir du cent cinquantième kilomètre. Il s'agit en somme d'un dispositif juste et efficace, en cohérence avec nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Si, sur ces dispositions, nous avons abouti à une position d'équilibre, il ne me semble pas opportun d'augmenter la fiscalité davantage. Il me paraît préférable d'accompagner

En effet, la modification de cette taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes est susceptible d'entraîner un risque indemnitaire de plusieurs centaines de millions d'euros pour l'État. Le seul effet de l'adoption de ces amendements serait de bouleverser cette taxe, qui permet aujourd'hui de financer de façon sécurisée l'Afitf.

Le transport routier de marchandises, qui représente 89 % des flux de marchandises dans notre pays et 6 % des émissions totales de gaz à effet de serre, doit s'engager sur la voie de la transition énergétique et réduire ses impacts, avec pour horizon la neutralité carbone en 2050. Dans la phase de transition des flottes de véhicules, avec l'arrivée progressive de motorisations à énergies alternatives, il nous faut trouver des solutions opérationnelles qui fournissent des résultats immédiats pour le bon suivi de cette trajectoire. La solution éco-combi apparaît comme pertinente dans le cadre de cette stratégie. Il s'agit d'une combinaison de deux remorques standardisées dont l'attelage permet une gestion simplifiée pour l'ensemble de la chaîne logistique- chargeurs, logisticiens, multimodal. Concrètement, un camion tracte deux semi-remorques au lieu d'une, soit deux fois plus de marchandises, c'est-à-dire 66 palettes au lieu de 33, pour un seul véhicule au lieu de deux. Avec cette solution, les trajets sont prédéterminés et impératifs, comme c'est déjà le cas pour les convois exceptionnels.

Les économies d'énergie réalisées doivent toutefois être rapportées à la tonne transportée. En effet, la consommation du véhicule augmente légèrement, de 8 % à 10 %, en fonction des usages et du poids tracté. Cet amendement vise donc à mener une expérimentation de deux ans en France, principalement sur les axes autoroutiers, de manière structurée et avec trois impératifs

Par ailleurs, au-delà des gains réalisés en matière de réduction des gaz à effets de serre et de compétitivité, il est nécessaire de prendre en compte dans cette expérimentation l'aspect sécuritaire. Ainsi, cet amendement vise également à assurer l'encadrement de cette expérimentation par le ministère des transports et le ministère de l'intérieur, particulièrement par la délégation à la sécurité routière. Je précise que cet amendement est issu d'un travail conjoint avec l'Union des entreprises de transport et logistique de France. Quel est l'avis de la commission ? Monsieur ? Monsieur le sénateur Redon-Sarrazy, il ne me paraît pas souhaitable de multiplier les dispositifs visant à augmenter la charge et la taille des véhicules de transport routier de marchandises.

le fond, plusieurs rapports ont déjà montré que les effets positifs allégués ne compensent pas les externalités négatives ; je pense à la dégradation des infrastructures, à l'impact en matière de sécurité routière ou encore simplement à l'acceptabilité sociale. Dès lors, plutôt qu'une approche théorique et générale, le Gouvernement a choisi d'expérimenter par voie réglementaire certaines dérogations, lorsqu'elles concernent un secteur d'activité mettant en avant des arguments qui lui sont spécifiques- le transport de betteraves, par exemple. En conséquence, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à modifier les obligations d'information instituées par le présent article pour promouvoir le recours aux biocarburants et à l'électromobilité.

les auteurs de l'amendement considèrent néanmoins que certains biocarburants, quand leur production n'entre pas de surcroît en concurrence avec des cultures vivrières, contribuent eux aussi à produire des émissions de gaz à effet de serre et n'offrent donc pas toujours un bon bilan carbone.

appliquerait cet objectif de 25 % à toutes les entreprises, ce qui ne me semble pas raisonnable au regard des différences importantes entre

ou encore à décarboner les nouvelles flottes de poids lourds, ont ainsi été adoptés en commission. Par ailleurs, il existe un risque important, vous le savez, que la mesure proposée ne soit particulièrement pénalisante pour nos concitoyens vivant en zone rurale, pour lesquels la livraison peut-être davantage nécessaire et sur lesquels il ne semble pas opportun de faire peser le coût

? Les auteurs de ces deux amendements posent une question importante : celle de l'impact de la livraison sur l'environnement. Ce sujet fait l'objet de travaux en cours. Je pense en particulier à la mission confiée à Anne-Marie Idrac, à Anne-Marie Jean et à Jean-Jacques Bolzan visant à proposer au Gouvernement une feuille de route en matière de logistique durable. savons que celle-ci est un maillon essentiel, qui peut contribuer à rendre la contribution environnementale du e-commerce neutre, voire positive. Il est également prévu que l'étude confiée à France Stratégie et à France Logistique, qui concerne les plateformes de e-commerce et l'immobilier logistique, approfondisse la question des modes rapides de livraison,

de livraison entre le dernier lieu de stockage et le domicile du client. Ce serait une manière vertueuse de favoriser l'implantation de zones de stockage

donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu'un point de retrait ou un établissement du fournisseur sont assujetties à une taxe forfaitaire en fonction d'un barème lié au montant de la commande. Ce dispositif vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre

commercialisent, le plus souvent à perte. C'est en partie ce qui explique qu'un géant comme Amazon dégage un résultat net aussi faible en proportion de son chiffre d'affaires- environ 1 %. Lorsque le législateur a interdit la livraison gratuite, les plateformes ont contourné le problème en proposant une livraison à quelques centimes. Au-delà des contraintes de concurrence déloyale qu'elles créent pour les commerces physiques, ces pratiques suscitent des flux de ce fait, des effets particulièrement préjudiciables en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de congestion routière, du fait des nombreuses rotations de véhicules. La crise sanitaire a démultiplié le nombre de livraisons de colis, corollaire de l'explosion du e-commerce.

et serait de nature à réduire l'empreinte carbone de la logistique de la livraison. Ainsi, une livraison le jour même pourrait être taxée à 3 % du montant de la commande, à 2 % à J+1 et à 1

Or la hausse des prix que vous proposez par ce dispositif peut être complètement disproportionnée par rapport au prix du produit qui est vendu. Deuxièmement, puisque cette taxe est proportionnelle à la distance, le dispositif pénalisera encore plus les consommateurs en zone rurale

Cette idée simple consiste à faire remonter le signal-prix au niveau du commanditaire de la prestation, sans que cela repose sur le transporteur, maillon faible de la chaîne Cette contribution est donc une incitation immédiate à utiliser des solutions de transport plus écoresponsables et permet de compléter l'ensemble des dispositions prévues et engagées pour le verdissement des flottes. disposition serait un signal favorable en faveur de la massification des flux de marchandises et contribuerait à replacer la chaîne logistique au centre du jeu, la volumétrie carbone étant très directement indexée sur la capacité des véhicules à circuler « à plein

en impliquant les secteurs les plus émetteurs dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ceux-ci devront rédiger des feuilles de route avec le Gouvernement et les collectivités locales visant à coordonner les actions mises en oeuvre par chacune des parties

Cet amendement vise à créer un label permettant de valoriser les entreprises de commerce en ligne engagées dans une démarche de logistique durable. Il s'agit de traduire la proposition n° 40 du rapport de la mission d'information relative au transport de marchandises et aux impératifs environnementaux. Quel est l'avis de la commission

Jean-Michel Houllegatte. Les auteurs de cet amendement, loin d'être opposés au tirage au sort pour favoriser l'implication des citoyens et citoyennes au sein des comités des partenaires créés par la loi d'orientation des mobilités, proposent de préciser la portée du dispositif. Ils souhaitent également demander au Gouvernement de réfléchir à la création d'un statut de « citoyen tiré au sort », qui favoriserait les réponses positives

habitants que l'ajout de citoyens tirés au sort ne remet pas en question la présence d'associations d'usagers ou d'habitants dans les comités de partenaires. En effet, les habitants tirés au sort ont potentiellement un intérêt plus large que ceux qui sont concernés par le projet. Par ailleurs, le

Le terme « intermodalité » renvoie à l'utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même trajet. Or aucun article de cette division ne favorise le recours à plusieurs modes de transport, notamment le train et l'avion, Dans un souci de clarté, nous pensons qu'il convient d'utiliser le terme adéquat et représentatif des dispositions de la division concernée. Nous considérons cependant que l'intermodalité est un enjeu central de la lutte contre le changement climatique pour favoriser le recours aux transports collectifs et à bas-carbone. Un plan d'action visant à développer l'intermodalité aux abords des gares et des aéroports est nécessaire. Il serait cohérent de l'inscrire dans le prolongement des aspirations de cette loi sur le climat. Ces dispositions ne figurent pas dans ce chapitre, et nous le regrettons.

derrière ce secteur littéralement à terre, du fait de la crise, il y a des hommes et des femmes, des usagers, une industrie et des emplois. Je ne participe pas non plus à ces critiques qui trouvent toutes vos propositions inacceptables. Les mesures sur l'aérien qui contribuent à l'effort de décarbonation ont de fortes conséquences. Nous avons la responsabilité de ne surtout pas fermer les yeux sur l'urgence, comme je l'ai entendu dire plusieurs fois aujourd'hui et comme le Groupe rappelé hier. Cette responsabilité implique de privilégier la voie du pragmatisme et de l'engagement et d'éviter que ce secteur ne fasse l'objet de nouvelles contraintes, même si le Gouvernement a pris en compte certaines remarques.

la taxe carbone, nous proposons d'adresser un message positif, tout en renvoyant le sujet à l'échelle de l'Union européenne pour ne pas créer un différentiel de compétitivité trop important. S'agissant des fameuses deux heures trente, les dispositions que nous avons clarifiées par la prise en compte des passagers en correspondance n'affecteront, dans les faits, qu'une ligne où le report modal est partiellement en cours. Nous proposons également de sanctuariser les lignes d'aménagement du territoire,

à préserver ces lignes d'aménagement du territoire. Nous proposons ainsi d'associer les collectivités locales aux décisions aéroportuaires et de réaménagement du trafic. Enfin, nous proposons une mesure

une définition juridique de la compensation carbone, qui serait ainsi la première en droit français, et nous proposons de séquestrer le CO2 en encourageant sa localisation en France ou en Europe. Pour conclure, nous préférons l'acceptabilité et le réalisme des mesures à l'interdit froid, qui a des effets plus cosmétiques qu'efficaces.

de ses propos. Cela mérite d'être souligné, parce qu'il n'est pas acceptable que le transport aérien soit montré du doigt comme il l'est, de manière souvent caricaturale, injuste et tout à fait disproportionnée.

cependant que les carburants alternatifs sont sans doute une solution plus pragmatique, qui sera opérationnelle à plus court terme, notamment pour les longs courriers.

en matière de gestion des plateformes aéroportuaires. Celles-ci sont en déséquilibre financier. Il revient aux collectivités de les remettre à l'équilibre, ce qui représente un coût important. La conséquence de cette stratégie dans une petite région comme la nôtre,

ne viendront pas remplacer la taxe de solidarité que nous devons au président Chirac. Madame la ministre, merci de nous confirmer que vous êtes d'accord avec la rédaction que nous proposons pour cet alinéa, sur ce point très précis. En effet, cela représente 400 millions d'euros

l'on a besoin de l'aérien, mais je suis également convaincu qu'il faudra que ce secteur paie le vrai prix de ses émissions de CO2 et que ce n'est pas 2 euros la tonne.

dont le secteur aérien devra s'acquitter à partir de 2025. Cet objectif devrait se traduire par un renchérissement structurel du coût des transports aériens. Il faut éviter que ce surenchérissement du coût des transports ne pénalise trop fortement les personnes les plus modestes, en particulier les personnes aux faibles ressources, qui sont plus nombreuses en outre-mer qu'en France hexagonale. Il est également nécessaire de protéger les étudiants, pour qui l'avion est l'unique moyen de transport reliant leur territoire avec l'Hexagone. Par

Cette proposition et, plus généralement, les débats qui ont déjà eu lieu et qui se poursuivent dans cet hémicycle au sujet de l'article 35 illustrent le caractère particulièrement clivant du transport aérien aujourd'hui. L'équilibre est difficile à trouver entre, d'un côté, la réduction des nuisances, et, de l'autre, le maintien de la continuité territoriale et de l'activité économique. Ce secteur Ce secteur est actuellement l'un des plus touchés par la crise sanitaire. Il n'est pas en mesure de faire face à une augmentation de sa fiscalité. Nous souhaitons donc utiliser ce temps pour réfléchir à la meilleure façon d'atteindre l'objectif que nous nous fixons en matière de prix du carbone préparer à mettre en place les instruments appropriés quand le secteur sortira de la crise. Le principe d'arrêter une surcote non documentée de 20 % par rapport au prix constaté sur le marché carbone pertinent ne paraît pas souhaitable. Mon avis est donc défavorable. 1687 rectifié, il est largement satisfait. En effet, dans la rédaction actuelle, l'article 35 prévoit que le rapport sur le prix du carbone prendra en compte un certain nombre d'enjeux, dont la continuité territoriale, qui est en fait la préoccupation sous-jacente à cet amendement, entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain. Cette question fera l'objet d'un examen spécifique dans le cadre du rapport. Je demande donc le retrait de

des mesures ont été prises. Cependant, comme cet article a une dimension programmatique, je veux rappeler que le Gouvernement, qui souhaite avancer vers la transition écologique du transport aérien, dispose d'un levier qu'il doit actionner de manière plus efficace. En deux mots, il s'agit de développer une gestion plus intégrée des vols dans leurs différentes phases de départ et d'arrivée, pour économiser du kérosène et du CO2. La

et à achever, sans retard supplémentaire, les grands programmes de modernisation de ce secteur. nous dressons le même constat que vous, ce qui prouve votre expertise en la matière. Les trajectoires vertes, ainsi qu'une optimisation des opérations aériennes au sol, peuvent réduire d'environ 10 % la consommation de carburant dans les émissions. L'aérien y travaille déjà,

Je partage le constat qui a été dressé : l'amélioration des opérations et de la performance opérationnelle peut vraiment contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. effet de serre. L'optimisation des routes aériennes constitue une ligne d'action constante de la direction des services de la navigation aérienne. Elle est partagée par les compagnies aériennes, qui y voient un levier pour réduire la consommation de carburant. Nous estimons, nous aussi, que l'amélioration des procédures de navigation aérienne pourrait réduire de 10 % à 15 % les émissions de l'aviation.

raison pour laquelle nous estimons nécessaire de réinstaurer le schéma national des infrastructures, qui permet de fixer les orientations de l'État en d'infrastructures et de services de transport ferroviaire relevant de sa compétence. Il est essentiel pour nos concitoyens d'avoir connaissance des objectifs de l'État en matière d'infrastructures, afin de faire face aux attentes sociales de mobilité et d'aménagement du territoire.

Il convient de réinstaurer ce schéma national, dont l'élaboration peut relever du Conseil d'orientation des infrastructures, qui a été institué par la LOM et qui doit être soumis à la validation du Parlement. détermine aussi, dans un souci d'aménagement et d'égalité des territoires, les services de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés par l'État qui répondent aux besoins de transport. Il s'agit des trains d'équilibre du territoire. Or il n'a jamais été élaboré. De plus,

Face à la politique de suppression des services de TGV sans correspondance mise en oeuvre par SNCF Voyageurs, il est urgent que l'État se saisisse de cette mission en présentant sa vision de la politique de dessertes nationales, le schéma national des services de transport.

Le scénario retenu au titre de la LOM présente l'intérêt, par rapport aux schémas antérieurs, de comporter de vrais choix stratégiques, desquels découle une réelle priorisation dans l'affectation des moyens.

Cependant, il ne me semble pas que la modification du rapport annexé à la LOM, créé il y a déjà deux ans, soit la meilleure manière de faire avancer les choses ; je parle sous le contrôle du rapporteur du projet son excellent rapporteur

madame la ministre, qui constitue bien une priorité de la LOM. Le Gouvernement a pleinement conscience de l'intérêt que présentent ces gares d'interconnexion pour faire le lien entre le transport de longue distance et les transports du quotidien. Mais la création de nouvelles

Afin de respecter nos objectifs climatiques, nous proposons que la France s'engage à mettre en place un véritable plan d'investissement en faveur du transport ferroviaire de voyageurs. D'ici à 2030, elle doit investir massivement dans la régénération du réseau ferré, sa modernisation et le renouvellement du matériel roulant. Ce plan d'investissement devra être mis en oeuvre dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi. Alors que la lutte contre le dérèglement climatique contraint à décarboner massivement le secteur des transports, premier émetteur de gaz à effet de serre, le train est un allié essentiel pour atteindre nos objectifs. le train est un mode de transport particulièrement performant d'un point de vue environnemental : il transporte 11 % de l'ensemble des passagers et 9 % des marchandises, mais il n'est responsable que de 0,3 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Il s'agit aussi d'un formidable outil d'aménagement du territoire, pourvoyeur de nombreux emplois non délocalisables. Le plan de soutien au transport ferroviaire, présenté par le Gouvernement en septembre 2020, marque une première étape importante, puisqu'il a permis de sécuriser les investissements prévus, malgré la crise sanitaire et économique. Ce plan est néanmoins insuffisant pour assurer une véritable relance de ce mode de transport. Nous considérons que ce plan d'investissement doit être considérablement renforcé. Il est en effet nécessaire d'investir 500 millions d'euros supplémentaires par an pour garantir une régénération satisfaisante du réseau structurant, 700 millions d'euros supplémentaires par an pour réussir la régénération des lignes de desserte fines du territoire, autrement dit des 200 millions d'euros supplémentaires par an pour réaliser l'ensemble des projets de modernisation et de développement du réseau identifié dans le scénario intermédiaire du rapport Duron et 150 millions d'euros supplémentaires par an pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et favoriser le développement d'un véritable réseau de trains de nuit en France et vers l'étranger.

importante, mais insuffisante pour garantir une régénération satisfaisante du réseau structurant et la régénération des lignes de desserte fine du territoire, pour réaliser l'ensemble des projets de modernisation et de développement du réseau identifié dans le scénario intermédiaire du rapport Duron et, enfin, pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et favoriser le développement d'un véritable réseau de trains de nuit. Je suis convaincu que cet amendement

n° 1530 rectifié vise la mise en place d'un plan d'investissement supplémentaire pour la relance du transport ferroviaire. Le principe en a déjà été acté dans la loi d'orientation des mobilités. Par ailleurs, le plan de relance comprend un volet ferroviaire de 5 milliards d'euros, montant qui s'ajoute à la reprise par l'État des 35 milliards d'euros de dette de SNCF Réseau. Ces contributions sans précédent de l'État vont permettre de financer la remise en état du réseau, de réaliser les aménagements nécessaires au développement du fret ou à la réouverture des lignes de trains de nuit. Je considère que, désormais, nous en sommes au stade de la mise en oeuvre des investissements, et non à l'élaboration

les lignes desservies par les TET sont indispensables à la desserte du territoire national. Elles offrent aux populations des zones les plus enclavées et les moins bien desservies une solution de mobilité pratique, rapide et écologique. s'agit aussi d'un outil contre la désertification des territoires ruraux et de développement. Le 14 juillet 2020, le Président de la République affirmait cette ambition en déclarant qu'il voulait développer le fret ferroviaire, les trains de nuit et les petites lignes de train. Il est temps de passer aux actes.

du rapport proposent notamment de rouvrir cinq lignes de jour, les lignes Bordeaux-Nice, Nantes-Rouen-Lille, Toulouse-Lyon, Metz-Lyon-Grenoble et Tours-Clermont-Ferrand-Paris, et de construire un véritable réseau de trains de nuit autour de quatre corridors, Bordeaux-Marseille,

Afin d'assurer le déploiement d'un tel réseau, cet amendement a pour objet que le Gouvernement présente au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un plan d'action qui détaille la façon dont il entend parvenir à cet objectif à l'horizon 2030. Nous demandons aussi que la commande de matériel roulant nécessaire pour atteindre cet objectif soit décidée avant la fin du premier semestre de 2022. En effet, il faut s'attendre à ce qu'un délai de cinq à sept ans sépare la prise de décision, c'est-à-dire la commande du matériel roulant, et la livraison.

Mme Béatrice Gosselin. Cet amendement tend à planifier le développement de l'offre de trains de nuit en direction des territoires touristiques français. En effet, les trains de nuit sont nécessaires au développement et au dynamisme des secteurs touristiques de notre pays. Ils constituent une solution de substitution moins coûteuse, notamment pour les familles et les jeunes, et permettent de réduire, de manière non négligeable, les déplacements carbonés.

Ainsi, les vols intérieurs en France, nécessaires pour désenclaver nos territoires, sont déjà soumis à de lourds prélèvements, avec en particulier des taxes d'aéroport, qui sont plus élevées chez nous qu'en Suède, par exemple, ce pays que vous aimez tant.

Cette mesure aurait un impact important sur l'attractivité de certains territoires et sur les citoyens, qui pourraient voir leur temps de trajet allongé, sans oublier la difficile identification des vols concernés.

La restriction du trafic aérien, en plus d'avoir de fortes conséquences économiques sur un secteur déjà fortement touché par la crise, viendra limiter la liberté du commerce et de l'industrie des transporteurs,

pénalisés par cette mesure.

Les vols en jet privé, aux tarifs inabordables pour une grande majorité de la population, ont des effets délétères sur l'environnement. Ils émettent dix fois plus de CO2 par personne que les liaisons aériennes commerciales, déjà très polluantes par rapport à d'autres modes de transport. En moyenne, un vol privé de quatre heures suscite autant d'émissions qu'un individu moyen en une année. D'ailleurs, entre 2005 et 2019, les émissions de CO2 des jets privés en Europe ont augmenté de près d'un tiers, soit plus rapidement que les émissions de l'aviation commerciale, et elles ont encore cru de façon exponentielle depuis la crise de la covid-19.

L'application de cette interdiction aurait aussi l'immense avantage d'encourager les constructeurs, les compagnies et les usagers à investir fortement dans la recherche et le développement en faveur de solutions durables et vertes pour ce mode de transport aérien.

dans ce cas, les vols ne sont pas couverts par le règlement européen concerné. L'extension de l'interdiction à ces vols remettrait fondamentalement en cause la liberté d'aller et venir. Ce serait comme interdire

est ancré dans l'organisation des territoires et des infrastructures. Le bruit ferroviaire illustre parfaitement les contradictions qu'il nous faut affronter. À cet égard, deux légitimités s'opposent souvent

le type de travaux visés par cet article, afin d'indiquer explicitement que l'interdiction de déclaration d'utilité publique, ou DUP, ne concernera que la création ou l'extension d'un aérodrome, d'une aérogare ou d'une piste d'atterrissage.

l'évaluation des émissions atmosphériques du secteur aérien. Les avions laissent sur leur passage des traînées de condensation, c'est-à-dire de petits nuages, dits cirrus, qui persistent pendant plusieurs heures. Si l'existence de ce phénomène est incontestable,

Dans le droit en vigueur et dans la pratique, les collectivités territoriales sont très attentives à la vie des aéroports lorsque leurs territoires sont concernés, qu'il s'agisse du développement local ou de la qualité de vie des riverains, des domaines de l'emploi, de la formation, de l'urbanisme, de l'environnement ou, bien sûr, des transports. Quel

fixer le socle législatif d'une compensation efficace en privilégiant les programmes de séquestration dans les puits de carbone situés notamment au sein de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

Personnellement, j'estime qu'il peut être quelque peu dangereux de se focaliser uniquement sur la France ou sur l'Europe.

de l'article 38, une priorisation des projets favorisant le renouvellement forestier, l'agroforesterie, l'agrosylvopastoralisme, le développement des prairies et de toute autre forme d'agriculture régénérative. Bien entendu, nous sommes favorables à cette précision. Nous souhaitons simplement apporter une clarification en direction de nos agriculteurs, car les pratiques agricoles ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre doivent également être prises en compte. Enfin, cet amendement vise à apporter une clarification rédactionnelle, en remplaçant la notion d'absorption du carbone par celle de compensation.

recours à la capture suivi de la séquestration ou de la réutilisation du CO2 à des fins de production de carburants synthétiques pour l'aviation. La captation, le stockage et le recyclage du CO2 sont en effet des technologies clés, qui nous permettront demain d'atteindre la neutralité carbone tout en bénéficiant de carburants à la fois propres et performants. Le présent texte doit ouvrir la voie

carbone » agricoles éligibles sur le marché de la compensation carbone des liaisons intérieures métropolitaines. La lutte contre le réchauffement climatique

pour lutter contre le changement climatique. Le label Bas-carbone, géré par le ministère de la transition écologique, garantit par ailleurs la qualité des crédits « carbone »

n'est pas limitative. En revanche, mentionner l'ensemble de l'agriculture semble ouvrir un périmètre un peu trop vaste. La

climat, à modifier le code de l'environnement afin d'intégrer dans le budget carbone de la France les émissions de gaz à effet de serre issues du transport aérien international. Le secteur aérien est la première source de croissance des émissions de CO2 en France ces dix dernières années,

La rénovation des bâtiments présente deux enjeux : un enjeu de pouvoir d'achat et un enjeu de décarbonation. Le logement est le premier poste de dépenses des ménages et il est la source de 27 % des émissions de CO2. Rénover des logements, c'est réduire les factures, lutter contre la précarité énergétique, relancer notre économie à travers l'activité du bâtiment et, au bout du compte, atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé d'un parc de logements basse consommation en 2050. Bien sûr, le défi est de taille : sur les 29 millions de résidences principales que compte notre pays, seulement 7 % sont déjà à ce standard, tandis que 17 % sont qualifiées de passoires thermiques.

Le texte de l'Assemblée nationale comporte des avancées : le renforcement de la lutte contre les passoires thermiques, la création d'accompagnateurs des ménages les plus modestes pour la rénovation, du prêt avance mutation garanti ou encore du plan pluriannuel de travaux. Pour autant, il était insatisfaisant. C'est pourquoi la commission des affaires économiques l'a enrichi, guidée par trois idées maîtresses : plus d'ambition, plus de solidarité, plus d'équilibre entre les nouvelles obligations et les nécessaires mesures d'accompagnement. L'ambition, c'est une définition cohérente de la rénovation performante et la prise en compte des logements de classe D. En effet, en 2050, le parc devrait être composé de logements de B, minoritairement de classe C, sauf exception. La solidarité, c'est, pour les ménages les plus modestes, un reste à charge minimal, la gratuité des accompagnateurs Sichel et la baisse de la TVA dans le logement social.

le secteur du bâtiment représente aujourd'hui 27 % des émissions de gaz à effet de serre en France. Les deux tiers de ces émissions sont issus du secteur résidentiel.

Or la grande majorité des propriétaires occupants sont des retraités ne percevant que de petits revenus. Il nous faut donc considérer cette réalité. Par voie d'amendements, le groupe Socialiste, Écologique et Républicain souhaite, de ce fait, promouvoir une véritable écologie sociale. Ses amendements ont pour objectif, en premier lieu, de prévoir une trajectoire plus ambitieuse de lutte contre les passoires thermiques en renforçant le niveau de performance à atteindre, en interdisant la location de tels biens à compter de 2030 et en contrôlant la qualité de l'exécution des travaux de rénovation. En second lieu, ils visent à renforcer les mesures de justice sociale, notamment en allant plus loin dans la prise en charge financière des ménages les plus modestes. L'ampleur du chantier visé est colossale et d'une grande complexité en raison des disparités territoriales. Or le projet de loi Climat et résilience, dépourvu d'étude d'impact, n'explicite que très peu, voire pas du tout, comment tous ces efforts seront financés. À cet égard, il nous semble indispensable de poser tout de suite certains préalables et de rétablir un équilibre entre écologie et justice sociale, afin qu'il n'y ait pas d'écologie à deux vitesses. La lutte contre le changement climatique ne peut pas bénéficier aux seuls ménages aisés. Dans ce combat, comme dans tous les autres, les plus modestes ne pourront pas pas être une fois de plus la variable d'ajustement. C'est une question d'équité face à un enjeu dont la gravité nous touche tous, sans exception. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas,

puisqu'il représente 26 % des émissions de gaz à effet de serre. Voilà qui explique parfaitement l'objectif, partagé, à la fois écologique et social d'en finir avec les passoires énergétiques : non seulement ces logements participent au dérèglement climatique, mais leurs

du fait des fourches caudines de l'article 40 de la Constitution, nous sommes extrêmement limités dans nos propositions. Ainsi, nous ne pouvons pas intervenir sur le reste à charge des opérations de rénovation, pas plus que sur les aides dont peuvent bénéficier les ménages en situation de précarité. Nous le regrettons.

D'ailleurs, sur l'ensemble de cette partie, la commission des affaires économiques a largement amélioré le projet de loi, en travaillant notamment sur l'idée d'un reste à charge minime pour les familles et en oeuvrant pour rehausser les objectifs de rénovation. En disposant des bons mots, nous traitons ainsi

IV intitulé « Se loger », titre ô combien structurant et central pour la mise en oeuvre des politiques de transition. En 2019, le secteur du bâtiment a émis 81 millions de tonnes de est donc le troisième secteur le plus émetteur derrière les transports et l'agriculture. Au-delà de la question centrale du climat, la massification des rénovations, qui doit clairement constituer une priorité nationale, permet de répondre aux enjeux en matière de relance économique, d'emploi, de santé publique et de pouvoir d'achat, grâce à la réduction de la facture d'énergie.

Il y va de l'efficacité des politiques publiques et de la parole donnée à la Convention citoyenne pour le climat, mais aussi du respect de nos engagements internationaux pour le climat. La stratégie du Gouvernement, qui consiste à déployer des politiques purement incitatives, à encourager les citoyens à rénover, à leur rythme, en espérant que les objectifs seront atteints en 2050, n'est malheureusement plus suffisante, comme le soutient également le Haut Conseil pour le climat. Il appartient au Parlement, et à vous, madame la ministre, de s'attaquer au gisement d'économies d'énergie considérables du bâti et de se retrousser les manches pour réussir le changement d'échelle attendu en la matière.

Il faut donc véritablement renforcer et davantage structurer le service public pour la performance énergétique des bâtiments à l'échelon local, de l'identification au suivi post-travaux. L'assistance à la maîtrise d'ouvrage doit être plus systématique en cas d'aide publique. La formation des artisans doit être renforcée. Pour atteindre 800 000 rénovations globales par an en rythme de croisière, et dans une logique de justice sociale, il est impératif d'apporter des moyens financiers suffisants pour subventionner intégralement des travaux de rénovation complets et efficaces, en priorité pour les ménages très modestes.

chers collègues, la précarité énergétique est un fléau : 15 millions de logements sont qualifiés de passoires thermiques, soit quelque 17 % des logements considérés comme très énergivores, catalogués F et G sur l'échelle de diagnostic de performance Les maisons individuelles, le parc privé ou ancien, les zones rurales et montagnardes, qui ont des besoins de chauffage importants, sont particulièrement concernés. À cet égard, la rénovation énergétique des logements fait partie intégrante de la politique écologique. indispensable pour respecter la trajectoire définie par l'accord de Paris, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, dont environ 25 % proviennent du logement. Conscients de ces enjeux, les Français plébiscitent le dispositif MaPrimeRénov'

les bâtiments », notre objectif est simple : accélérer la rénovation énergétique de nos logements, en massifiant et en accompagnant de façon efficace tous les travaux de rénovation, de façon juste, en portant attention aux plus fragiles.

le gel de l'augmentation des loyers de ces logements d'ici à 2028 ; la mise en place d'outils d'évaluation- le DPE, l'audit, le diagnostic technique global -, du plan pluriannuel de travaux, du prêt avance mutation- il permettra de financer le reste à charge, y compris pour les ménages ayant difficilement accès au crédit classique -et d'un accompagnement de confiance pour tous les ménages, conformément aux recommandations de la mission Sichel.

porte sur la définition de la rénovation performante. Cette question arrivera dans le débat et il me semble important d'adopter une définition pragmatique, réaliste, qui permette de porter le parc en moyenne autour de l'étiquette B, c'est-à-dire A, B ou C, à l'horizon 2050.

économiques ? Prévoir que le contenu du diagnostic de performance énergétique doit être exprimé en énergie finale serait contraire au droit de l'Union européenne. En effet, la directive européenne du 30 mai 2018 sur la performance énergétique des bâtiments, issue du paquet d'hiver européen,

un classement spécifique et adapté au climat des outre-mer, au regard de la notion de confort thermique différencié qui les caractérise et des inégalités de traitement auxquelles ces territoires seraient soumis si le classement hexagonal leur était appliqué en l'état. Les nouveaux DPE s'appuient sur les seuils de performance énergétique et les composants de la construction. Or la méthode de calcul permettant de définir la performance énergétique d'un logement ou d'un bâtiment s'appuie en outre sur le « coefficient de rigueur climatique donné par la répartition des zones climatiques en France. Ce zonage, élaboré avec le concours de Météo France, détermine huit zones climatiques en fonction des températures en période hivernale et en fonction des températures estivales. Il exclut les outre-mer, alors même que ces zones climatiques permettent d'optimiser les normes de construction en fonction des territoires. De même, il convient de préciser que le confort thermique de l'Hexagone est différent de celui des territoires des outre-mer. Il y a donc lieu de différencier nos politiques, à la fois pour la métropole et pour les outre-mer. Quel

un classement général dont les modalités d'application seront précisées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Dans cet amendement, il est fait référence aux zones climatiques et d'altitude et de confort thermique. Celles-ci sont définies par l'article R.

a déjà été pris en compte dans le projet de loi. Ainsi, l'article 39 intègre cette notion à la définition de rénovation énergétique performante et l'article 39 prévoit

M. Daniel Salmon. La rénovation des bâtiments tertiaires constitue un axe majeur de décarbonation. Le tertiaire représente en effet 42 % des émissions du secteur du bâtiment. Cet amendement vise à répondre à la demande de la Convention citoyenne pour le climat de contraindre les espaces publics et les bâtiments tertiaires à réduire leur consommation d'énergie. son objet les objectifs du décret tertiaire, en contraignant ces bâtiments à réduire leur consommation d'énergie et en renforçant l'obligation de rénovation thermique, il tend à établir une obligation de résultat, et non de moyens, et à fixer une valeur à atteindre et non une démarche à entreprendre. Les propriétaires ont donc la liberté de décider des moyens à mettre en place, du moment que l'objectif est atteint.

Il précise qu'une trajectoire d'obligation de rénovation, exprimée en termes de performances énergétiques et climatiques, pourrait inclure l'ensemble des bâtiments tertiaires, conformément aux objectifs de la

Varaillas. Cet amendement vise à répondre à la demande de la Convention citoyenne pour le climat de contraindre, par des mesures fortes, les espaces publics et les bâtiments tertiaires à réduire leur consommation d'énergie, en dehors des obligations pesant sur les seules collectivités, comme c'est d'ailleurs prévu à l'article 39. En effet, la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment doit mobiliser l'ensemble des acteurs. Nous estimons ainsi que les locaux professionnels et publics, peu importe d'ailleurs leurs propriétaires, doivent être soumis à des obligations de performance énergétique. Nous proposons, par conséquent, de renforcer l'obligation de rénovation thermique de l'ensemble des bâtiments du secteur tertiaire en fixant une trajectoire d'ici à 2060. Par ailleurs, nous proposons de réintroduire la distinction entre consommation d'énergie finale et consommation d'énergie primaire, ainsi que la référence à la consommation de l'ensemble du parc en valeur absolue. Leur suppression dans la loi ÉLAN a introduit des marges d'interprétation très importantes, qui constituent un recul par rapport aux textes préexistants.

ces objectifs, dès lors qu'ils sont exprimés en énergie finale, peuvent aboutir au remplacement de systèmes de chauffage utilisant les énergies renouvelables- je pense par exemple aux réseaux de chaleur -par des systèmes de chauffage électrique, sans amélioration de la performance environnementale du bâtiment. Cet amendement vise donc à exprimer les objectifs de réduction de de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires également en énergie primaire, afin de prendre en compte la chaleur perdue, laquelle peut atteindre deux tiers lors de la conversion en énergie électrique. Cela permettrait également d'encourager les maîtres d'ouvrage à recourir à une solution globale de rénovation énergétique et à réaliser des efforts sur l'enveloppe du bâtiment, afin de réduire les besoins en énergie de l'ensemble des usages du bâtiment. La parole est à M. Guy Benarroche,

jusqu'à 60 % de leur consommation d'énergie d'ici à 2050 par une obligation de rénovation de certains d'entre eux. À mon sens, cela poserait

toute référence aux actions, qui peuvent englober- je vous le rappelle -la mise en place d'un système de management de l'énergie, l'autoconsommation de la chaleur fatale produite par le bâtiment ou encore une régulation fine de leurs fournitures

bâtiments tertiaires, par ailleurs non précisément définis, alors que l'ensemble d'entre eux sont actuellement concernés. Les auteurs

primaire en plus de l'énergie finale dans les objectifs de réduction de la consommation d'énergie des bâtiments tertiaires. Cette modification me semble tout à fait dispensable. En effet, l'objectif global de réduction de 50 % de notre consommation d'énergie d'ici à 2050 figurant à l'article L. 100-4 du code de l'énergie est exprimé en énergie finale.

bâtiments publics. L'État et les collectivités territoriales et leurs groupements auraient ainsi la possibilité de recourir à un financement différé de leurs travaux de rénovation énergétique. Certes, de telles règles sont très encadrées par le droit de l'Union il est très utile de pouvoir les faire évoluer pour rénover pleinement et effectivement notre parc de bâtiments publics. Aussi les souplesses administratives proposées dans ces deux amendements identiques doivent-elles être accueillies positivement. J'émets donc un avis favorable sur ces deux amendements

Pour le Conseil constitutionnel, l'interdiction du paiement différé fait partie des règles de droit commun de la commande publique auxquelles il ne peut être dérogé qu'avec prudence, afin de ne pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics. C'est pourquoi le préfinancement est réservé aux marchés de partenariat, qui sont plus strictement encadrés, compte tenu de leur caractère dérogatoire de droit commun aux marchés publics. L'adoption des amendements présentés aurait pour effet d'abolir la distinction entre les contrats globaux et les marchés de partenariat, niant le caractère dérogatoire et sensible du préfinancement et contournant l'encadrement propre à ces contrats imposé par le Conseil constitutionnel.

la prise en compte de l'impact carbone sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, y compris durant ses phases de construction et de démolition. Cela va entraîner une transformation profonde des types de bâtiments et modes de construction, notamment du fait de la disparition progressive du chauffage exclusivement au gaz et de la montée en puissance rapide des systèmes constructifs bas-carbone, notamment bois et

objectifs. Ainsi, les normes applicables aux logements individuels, aux logements sociaux ou aux réseaux de chaleur seront de plus en plus exigeantes à compter de 2022. C'est nécessaire

permet de déployer une stratégie qui dépend en grande partie des informations en matière de consommation énergétique. Celles-ci sont données par de tels outils et sont à la portée des administrateurs à l'échelle nationale et locale. Le diagnostic calcule précisément la consommation énergétique des logements, ainsi que leurs émissions de gaz à effet de serre. Le Haut Conseil pour le climat, dans une lettre datée du 22 mars 2021 adressée au ministère de la transition écologique, déplore les paramètres utilisés dans le calcul du diagnostic de performance énergétique,

qui apprécie l'énergie réellement consommée dans la nature, et don la méthode de calcul est controversée. Par exemple, le facteur d'émission de CO2 du chauffage électrique, qui permet de détailler le contenu gaz à effet de serre, est passé

Aussi, au vu des divergences sur les méthodes de calcul du diagnostic de performance énergétique, dans un souci de transparence et de recherche d'efficacité, il conviendrait de soumettre les paramètres techniques et les méthodes de calcul à l'avis indépendant du Haut Conseil, qui les encadrerait ainsi. Comme je l'ai

D'abord, les différents documents réglementaires, au premier rang desquels le DPE, ont été soumis, pour consultation, au Conseil supérieur de l'énergie, au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et au public. Ensuite, le Haut Conseil pour le climat, dont les effectifs- c'est un constat -sont tout de même très resserrés, et dont le profil est plutôt généraliste, peut de toute manière déjà être saisi par le président de chaque assemblée ou traiter de toute question relevant de sa compétence, y compris

comme les pompes à chaleur ne sont pas adaptés à tous les logements. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à lutter contre la précarité énergétique en demandant au Gouvernement de prendre des mesures mesures permettant d'accélérer le remplacement des anciens convecteurs électriques dans les logements considérés comme des passoires thermiques. Quel est l'avis de la commission

D'abord, les aides budgétaires ou fiscales existantes en matière de rénovation énergétique n'excluent pas du tout ce type de renouvellement. Ensuite, l'effort de renouvellement des systèmes de chauffage ne doit pas être limité à l'électricité. Il y a aussi le gaz

Compte tenu du rythme des innovations en matière d'efficacité énergétique, la méthode de calcul qui a été remise à jour deviendra insuffisante, voire obsolète, dès qu'il y aura de nouvelles avancées technologiques. Il est donc nécessaire de prévoir une remise à niveau régulière de la méthode de calcul du DPE,

approche de la rénovation thermique des bâtiments doit être engagée afin d'éliminer les passoires thermiques en dix ans et de sortir 12 millions de personnes de la précarité énergétique. Il faut prioriser les logements les plus énergivores et- c'est essentiel -préfinancer jusqu'à 100 % des coûts de la rénovation thermique pour les ménages les plus modestes. Le projet de loi prévoit la mise en oeuvre d'un système d'aides publiques et un reste à charge financièrement soutenable et incitatif pour les ménages les plus précaires. Le financement des travaux de rénovation est un frein majeur. Les montants de travaux sont élevés, de l'ordre de 300 euros à 400 euros en moyenne par mètre carré pour une rénovation globale, et les restes à charge seront difficilement supportables pour les plus modestes. Il est donc essentiel de préfinancer les coûts de rénovation en fonction des ressources des ménages. Constitution nous empêche d'être plus précis sur ce point, mais c'est bien un reste à charge équivalent à zéro qu'il faudra proposer à certains ménages. Notre amendement vise donc à garantir un reste à charge financièrement soutenable aux ménages modestes. C'est un préalable pour atteindre les objectifs de rénovation de la France, mais c'est aussi une exigence

d'un reste à charge financièrement soutenable et incitatif pour les bénéficiaires les plus modestes. Cet amendement tend à modifier la rédaction du texte afin de réellement garantir ce reste à charge, en substituant le terme « garantit » au terme « vise Cela nous permettra d'atteindre nos objectifs en matière de rénovation performante des habitations, nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique, et, surtout, de le faire de manière égalitaire, en soutenant les ménages précaires et en favorisant les travaux les plus ambitieux.

de l'accès aux aides, modulées en fonction des conditions de ressources, à la prévention de tout effet de bord financier négatif de la nouvelle définition de la rénovation énergétique performante et, enfin, à l'évaluation des conséquences financières de ces évolutions

Il peut en effet exister des cas d'équipement ou de rénovation très coûteux, pour lesquels l'État ne peut pas garantir une prise en charge complète, y compris pour les ménages modestes. À titre d'exemple, s'il est légitime de demander à l'État un reste à charge minimal sur certains équipements de première nécessité,

L'objectif du présent projet de loi de mettre fin aux passoires thermiques implique notamment la rénovation de 1,2 million de logements en location. Les propriétaires de ces logements devront financer plus de 13 milliards de travaux de rénovation énergétique pour ne pas tomber sous le coup de l'interdiction progressive de mise en location des passoires thermiques. Il convient toutefois de mieux prendre en considération le cas des logements mis en location, plus particulièrement ceux qui sont loués pour un prix modeste. Le coût des travaux de rénovation ne pourra ni être financé par les loyers tirés de la location du logement ni être compensé par les économies d'énergie générées par la rénovation, qui bénéficieront au locataire. Les aides proposées sont par ailleurs bien souvent insuffisantes pour permettre à ces propriétaires bailleurs, souvent de petits propriétaires, d'effectuer ces rénovations énergétiques. Aussi, le présent amendement tend à prévoir que les dispositifs de soutien à la rénovation énergétique devront aider ces propriétaires et prendre en compte le montant des loyers appliqués par ces derniers. Quel

est à Mme Viviane Artigalas. La loi devra fixer les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment pour deux périodes successives de cinq de cinq ans, en cohérence avec l'objectif de disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments basse consommation aux normes. La loi évaluera également le rythme et la

contre 46 % dans le Cantal, par exemple. Cette disparité s'explique par le fait que les typologies d'habitation et les conditions climatiques peuvent être très différentes d'un territoire à un autre. Les techniques et l'intensité de la rénovation énergétique potentiellement réalisable doivent donc pouvoir être adaptées. Notre amendement vise ainsi à proposer que le rythme et la typologie des rénovations nécessaires à l'atteinte des objectifs de rénovation prennent en compte les spécificités de chaque territoire.

que, dans le cadre de la loi quinquennale, à compter de 2023, le législateur détermine lui-même un rythme de rénovation selon une typologie précise- gestes de travaux, bouquets de travaux, rénovations globales ou performantes. L'amendement proposé

concernant les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment à l'horizon 2050, afin de disposer d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L'un des moyens proposés pour atteindre ces objectifs est d'inciter les entreprises artisanales du bâtiment à se réunir dans des groupements momentanés d'entreprises (GME), afin de favoriser la massification des travaux. Il peut s'agir par exemple de l'extension d'un bâtiment, de l'amélioration de la performance énergétique d'une maison individuelle,

les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment souhaitent avoir un interlocuteur unique, véritable facilitateur, dès lors qu'ils envisagent des travaux de rénovation énergétique

à 100 000 euros hors taxes, en permettant la mention de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client maître d'ouvrage, sauf si ce dernier l'exige.

prévue par l'article L. 124-3 du code de la construction et de l'habitation, à titre d'exception. Ces amendements visent à faire en sorte qu'elle devienne la règle, sauf demande du client. Ils opèrent donc un renversement de priorité sans véritablement changer le droit en vigueur. Cette observation faite, je reconnais qu'il est souhaitable de favoriser le développement des groupements momentanés d'entreprises pour faciliter les opérations de rénovation globale

Catherine Procaccia. Cet amendement vise à recentrer l'objectif défini à l'article L. 100-4 du code de l'énergie sur les classes de performance A ou B, au sens du nouvel article L. 173-1-1 du code de la construction

En appui de ces objectifs ainsi reformulés, le label BBC Rénovation pourra être recentré par voie réglementaire sur l'atteinte de la classe B ou A. Quel est l'avis de la commission

est une ambition louable sur le principe, mais son impact sera lourd. Il conduit non seulement à discriminer le gaz renouvelable, mais aussi à restreindre les choix des consommateurs,

revenir à la définition de la rénovation performante proposée par le Gouvernement et adoptée à l'Assemblée nationale. Cette définition prévoyait plusieurs critères cumulatifs : le gain d'au moins deux classes de DPE, l'étude de six postes de travaux de rénovation et l'atteinte de la classe A, B ou C. Le texte issu de la commission du Sénat prévoit de restreindre ce dernier critère à l'atteinte de la classe A ou B. En visant uniquement ces deux classes, vous demandez un niveau de performance très exigeant, alors que l'atteinte de l'étiquette C du DPE pour une partie des bâtiments existants

Par ailleurs, atteindre l'étiquette A ou B peut être impossible dans de nombreux cas, pour diverses raisons architecturales, patrimoniales ou économiques. Les conditions de dérogation à l'atteinte de ce niveau minimal restent drastiques, puisqu'il faut avoir intégralement traité les six postes de travaux. Si nous voulons inciter un maximum de ménages à engager des rénovations performantes, il semble préférable de qualifier de performantes un spectre un peu plus large de rénovations.

Mme Annick Billon. L'article 39 introduit la définition d'une rénovation performante dans le code de la construction et de l'habitation, cette définition ayant vocation à servir de référence pour les dispositifs d'aide à la rénovation énergétique. Il prévoit des critères plus souples pour les logements caractérisés par des particularités techniques, architecturales ou patrimoniales ou pour lesquels le coût des travaux pour atteindre une rénovation dite « performante » serait manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

à ajuster les délais pour la rénovation globale et à réécrire la référence à la qualité de l'air pour la rénovation performante. L'amendement que vous proposez, s'il était adopté, introduirait de fait un nouveau critère

En effet, la priorité est de permettre l'étalement dans le temps du bouquet de travaux pour que la rénovation soit soutenable financièrement.

Il est ainsi proposé de favoriser des rénovations qui permettent d'atteindre des objectifs ambitieux, en regroupant les interventions sur les différents postes de travaux dans une temporalité courte, c'est-à-dire dix-huit

accompagné par un opérateur de l'État, les travaux de rénovation puissent être réalisés par tranches, dans un délai maximum de six ans et à partir du moment où la totalité des travaux a été prévue. S'il est évident que des travaux réalisés en une seule fois permettent d'assurer une efficacité maximum, il est tout aussi important d'être en mesure de proposer un parcours de réhabilitation qui soit soutenable financièrement et supportable en site occupé.

Cela me semble contrevenir à deux principes qui ont guidé les travaux de la commission des affaires économiques : l'ambition de l'objectif et la simplification du dispositif.

me semble-t-il, à un besoin de souplesse demandé par tous les acteurs, que ce soit les professionnels de la construction ou ceux de l'énergie, mais également les associations de protection de l'environnement, monsieur Salmon. De plus, tel qu'il est rédigé, l'amendement tend à réintroduire une référence à la rénovation énergétique complète, ce contreviendrait à la position de notre commission, qui a souhaité supprimer cette catégorie dans un souci de simplification- nous avons répondu en cela à une demande formulée là aussi

amendement conduirait à retirer de la souplesse au dispositif, qui constitue pourtant, nous semble-t-il, le meilleur gage de son acceptabilité et de son applicabilité.

à prévoir une réalisation par tranches jusqu'à six ans lorsqu'une rénovation énergétique globale est réalisée par un propriétaire occupant. Si des ajustements

de l'article 39 permet déjà de déroger à un certain nombre de critères en cas de contraintes techniques, architecturales, patrimoniales ou économiques. L'objectif de ces amendements est donc assez largement satisfait.

leurs établissements publics et leurs groupements à recourir à un tiers investisseur pour financer les travaux énergétiques de leurs bâtiments, ce que le code de la commande publique ne permet pas pas actuellement. Il vise ainsi à lever un frein budgétaire à la rénovation énergétique des bâtiments publics et à mettre en oeuvre une nouvelle solution de financement pour l'État et les collectivités territoriales.

aux voix l'article 39. ter J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est parvenue à l'adoption d'un texte commun.